La procédure accélérée a été engagée sur ces textes.

Monsieur le président, messieurs les ministres d’État, mes chers collègues, comme dans la société tout entière, la lutte contre le trafic de stupéfiants a réuni un large consensus au sein de notre assemblée.

Nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers et nos magistrats combattent ce fléau depuis longtemps. Notre pays se trouve désormais à un point de bascule. Si nous ne réagissons pas avec fermeté et célérité, nous pourrions bien être dépassés par ce défi. Pour lutter efficacement, nous devons avant tout changer de regard sur les stupéfiants. Trop longtemps, les expressions « drogue douce » ou « usage récréatif » ont occulté la réalité tragique du terrain. Alors que l’on compte plus de 1 million de consommateurs de cocaïne dans notre pays, les stupéfiants sont devenus un marché très juteux, qui pourrait représenter 6 milliards d’euros. Avec de tels montants en jeu, les délinquants ne reculent devant aucune forme de violence. Dans certaines zones de la République, les contrôles d’identité et les fouilles sont menés non plus par les forces de l’ordre, mais par les trafiquants eux mêmes.

La rentabilité des trafics permet aux délinquants d’investir dans du matériel et des technologies avancées, ce qui rend d’autant plus difficile le travail des forces de l’ordre. Tout cet argent doit ensuite être blanchi, ce qui implique le développement de nombreuses ramifications au sein de notre économie. Les stupéfiants ne constituent bien souvent qu’un pan parmi d’autres de l’activité des réseaux de la criminalité organisée. Cela explique et justifie le choix de créer un parquet spécialisé dans ces affaires,

Ils minent le développement de nos territoires et empoisonnent la vie de nos concitoyens. Dans la droite ligne des récentes opérations « place nette », nous devons poursuivre nos efforts. Lors de nos débats, nous avons enrichi le texte de nombreuses mesures. Nous avons ainsi sécurisé les dispositifs de fermeture administrative des lieux Le Sénat a par ailleurs interdit le paiement en espèces des locations de voiture. Cette mesure permettra de lutter contre le blanchiment en favorisant l’identification des loueurs. Plusieurs amendements ont assujetti de nouveaux acteurs économiques aux dispositions de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Grâce à l’adoption d’un amendement de notre collègue Pierre Jean Rochette, les confiscations de véhicules seront désormais automatiques, y compris lorsque ceux ci sont immatriculés à l’étranger. Le Sénat a également accepté de mieux protéger les interprètes, acteurs clés de nombre de procédures, en adoptant un amendement de notre collègue Louis Vogel. Lorsque cela sera nécessaire, l’interprète pourra être autorisé par le magistrat à conserver l’anonymat. Sortir la France du piège du narcotrafic est un objectif nécessaire et ambitieux. À cet égard, nous pouvons regretter que le présent texte soit une proposition de loi et non un projet de loi. Le droit pénal et la procédure pénale emportent de lourdes conséquences sur les libertés de nos concitoyens. Il va sans dire que le travail de la commission des lois du Sénat est de grande qualité. Cependant, disposer d’une étude d’impact et de l’avis du Conseil d’État aurait sans doute permis de conforter la solidité juridique de plusieurs dispositions. La navette devra continuer d’améliorer le texte. Renforcer notre arsenal ne suffit pas. Pour gagner ce combat, nous avons également besoin de l’engagement de la justice et de nos services d’enquête. Les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires tiennent à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui luttent au quotidien contre ce fléau. Le projet de regrouper les cent plus gros trafiquants dans une prison de haute sécurité paraît nécessaire pour priver effectivement les réseaux de leurs chefs. Il met cependant en lumière le manque de moyens de la pénitentiaire : il nous faut à la fois construire davantage de places de prison et moderniser nos établissements.

nous ne pouvions en débattre. Nous considérons cependant qu’il est aussi commode que fallacieux de prétendre, comme le font certains de nos collègues, que le trafic de stupéfiants est une conséquence de l’économie de marché. de l’économie de marché. Les mêmes prônent la dépénalisation et l’augmentation des aides sociales pour lutter contre la criminalité : cela pourrait prêter à sourire si cet angélisme ne bénéficiait pas au développement des cartels.

Les centaines de victimes assassinées, parfois dans des conditions atroces, ont subi ce sort pour que la drogue parvienne au consommateur. Personne ne peut plus ignorer

ce que nous avions prévu pour le terrorisme, d’un parquet national anti criminalité organisée (Pnaco). Au delà du trafic de stupéfiants, c’est une criminalité totale qui est organisée.

nous devons nous prononcer aujourd’hui sur une proposition de loi à l’intitulé ambitieux : « sortir la France du piège du narcotrafic ». Ce texte s’est nourri des travaux de la commission d’enquête dont j’ai été vice présidente. nous avons dressé un état des lieux très préoccupant de ce phénomène, qui, d’année en année, gagne en ampleur et s’étend sur l’intégralité du territoire national, jusqu’à toucher nos petites villes et nos campagnes. Personne n’est épargné. Face à l’urgence, Étienne Blanc et Jérôme Durain, respectivement rapporteur et président de cette commission d’enquête, ont décidé de déposer cette proposition de loi. Ce texte, j’y insiste, est très ambitieux, en ce qu’il vise à renforcer les moyens procéduraux dans la lutte contre le narcotrafic. Les travaux de la commission d’enquête ont clairement démontré que nous accusions un retard considérable par rapport aux trafiquants. Ces derniers ne manquent ni de moyens ni d’imagination pour contourner les règles en vigueur et importer et vendre leur marchandise.

tant par les sénateurs que par le Gouvernement. Pour moi, ce sont des avancées décisives dans la lutte contre le narcotrafic. Il en va de même des dispositions qui visent à frapper les narcotrafiquants au portefeuille afin de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent. C’était l’une des recommandations phares de la commission d’enquête. Ainsi, je salue les mesures prévues aux articles 5 et 5 , qui permettront, au travers d’un mécanisme judiciaire ou administratif, de geler les avoirs des trafiquants. Vous le savez, ces individus n’ont aucune limite. Nous connaissons la dangerosité de leurs méthodes et de leurs moyens. J’ai une pensée émue pour les familles des deux agents pénitentiaires

Notre collègue Étienne Blanc a d’ailleurs proposé un dispositif complémentaire pour les appareils mobiles. Ces méthodes constituent un ajout pertinent aux techniques d’enquête existantes. Si nous pouvons nous féliciter d’avoir élaboré un texte très riche, nous devons admettre que des failles persistent. Je pense notamment à la prévention, volet pourtant primordial à mes yeux, qui n’a pas eu droit de cité dans cette proposition de loi. Je regrette que l’amendement que j’ai introduit à cet égard n’ait pas obtenu l’approbation de la commission des lois. Beaucoup d’entre vous m’ont affirmé que ce n’était ni le lieu ni le moment d’aborder cette problématique. Alors, dites moi : quand allons nous le faire ? Je ne doute pas une seconde que ce texte permettra de lutter efficacement contre le narcotrafic. Mais, il faut l’admettre, ses effets se concentreront essentiellement sur le haut du spectre.

L’an passé, le voyage s’est interrompu aux portes de l’aéroport guyanais pour plus de 1 000 mules en quête d’argent facile. Ce ne doit plus être une fatalité. Au delà de cette proposition de loi, il est primordial de mettre en place des actions pour endiguer le phénomène des mules, qui frappe de plein fouet les territoires ultramarins. Je pense notamment à un scanner corporel capable de détecter les objets ingérés. Messieurs les ministres, il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez vous. Monsieur le ministre de l’intérieur, votre prédécesseur, ici présent, s’était montré favorable, devant la commission d’enquête, à l’installation de scanners aux aéroports parisiens, points d’arrivée des vols en provenance de Guyane et des Antilles. J’espère que vous ferez toujours de ce dossier une priorité. Le scanner a fait ses preuves à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol aux Pays Bas. Je reste convaincue, tout comme l’ensemble des parlementaires ultramarins, que cette mesure peut endiguer ce phénomène dans nos territoires. Elle permettra, par la même occasion,

et d’Étienne Blanc, auteur de ce texte. Le groupe RDPI avait souscrit aux conclusions de la commission d’enquête ; il est donc tout à fait naturel qu’il soutienne aujourd’hui les objectifs de ce texte. Notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi.

a mis en lumière des phénomènes tels que l’ubérisation du trafic, l’extension du narcotrafic aux zones rurales ou encore la banalisation des drogues dures. Le texte que nous allons voter est le résultat à la fois du travail de cette commission d’enquête, de celui réalisé ensuite par les rapporteurs de la commission des lois et, de manière plus originale, des apports nombreux du Gouvernement, qui a su se saisir de ce véhicule législatif pour en renforcer la pertinence.

cette proposition de loi n’est pas un petit texte. Elle est, au contraire, absolument majeure. Voilà quelques années, notre procédure pénale était relativement uniforme. L’évolution de la lutte contre le terrorisme a modifié cet état de fait et nous avons commencé à voter des prérogatives exceptionnelles, car l’urgence et la matière le commandaient. Sur bien des aspects, nous nous apprêtons à élargir les exceptions conçues pour le terrorisme à la lutte contre le narcotrafic. C’est un fait. Tel est le choix, souverain, de cette assemblée. À la lecture du rapport de la commission d’enquête, il s’agit même d’un choix nécessaire, tant le narcotrafic se répand de manière incontrôlée dans l’Hexagone et dans nos territoires d’outre mer. Un pourcentage à lui seul est tout à fait édifiant : 80 % à 90 % du nombre total des règlements de compte s’expliquent par des différends liés au trafic de stupéfiants. Les conséquences en matière de santé publique sont également dramatiques. Les chiffres relatifs à la consommation de cocaïne ont été rappelés. par ce produit, le marché américain se tournant de plus en plus vers les drogues de synthèse. Qui plus est, ce texte est attendu, tant par les services de police que par les magistrats, qui ont besoin d’une plus grande coordination et des outils que nous allons leur offrir pour mener à bien leur travail avec plus d’efficacité.

la possibilité de fermer administrativement les lieux soupçonnés de blanchiment d’argent, la systématisation des enquêtes patrimoniales ou encore la création d’une interdiction administrative de paraître et la facilitation de l’expulsion des logements sociaux. Ces dernières mesures ne figuraient pas dans les préconisations de la commission d’enquête. Les services d’enquête apprécieront particulièrement l’amélioration de la coopération avec les services de renseignement et l’expérimentation du renseignement algorithmique, l’accès facilité aux messageries cryptées, le renforcement des outils à disposition des agents infiltrés, l’extension du régime des repentis et des mesures pour éviter que les trafiquants ne continuent de gérer leurs affaires depuis leur centre La procédure pénale sera nettement modifiée avec la prolongation de la garde à vue des mules, la fin du plafonnement des peines applicables aux infractions réalisées concomitamment, la création d’un « dossier coffre permettant de ne pas soumettre des pièces de la procédure et des techniques d’investigation au contradictoire et enfin la refonte du régime des nullités, dont il ne semble pas inutile de rappeler qu’elles sont uniquement soulevées par les avocats et non provoquées. Toutes ces mesures, nombreuses, sont substantielles. Un grand radical, Clemenceau, a dit un jour à cette tribune : « Le Gouvernement a pour mission de faire que les bons citoyens soient tranquilles, que les mauvais ne le soient pas. » De ce point de vue, nul doute que ce texte atteint cet objectif. Clemenceau avait tout de même ajouté : « […] et que les hésitants, que ceux qui ne savent pas, trouvent un point d’appui dans la loi C’est précisément sur ce point que je veux insister. Nous nous apprêtons à confier des prérogatives très importantes à nos services de police et de justice. Cela témoigne de la grande confiance que leur accorde notre assemblée. Est il besoin de rappeler qu’avec plus de pouvoir viennent plus de responsabilités ? Toutes ces techniques et dérogations n’ont qu’une seule fin : la lutte contre le narcotrafic. Aussi resterons nous attentifs à leur utilisation. De même, certaines mesures, à notre sens, demeurent perfectibles. Nous comptons sur la suite de la navette pour parvenir, notamment,

Quant aux « hésitants » de Clemenceau, ils existent. Ce texte, dont je comprends que ce n’est pas l’ambition, ne s’intéresse pas à eux. En dehors d’une mesure visant à dissuader le recrutement des plus jeunes par les réseaux, aucun dispositif de prévention n’est prévu. Or il faut garder à l’esprit que le narcotrafic tend à structurer l’espace social. Nous avons beaucoup parlé de l’Amérique latine au cours de l’examen de ce texte et du risque de « mexicanisation » auquel nous sommes vraisemblablement confrontés. Mais l’extension du narcotrafic sur ce continent n’est pas simplement liée aux outils qui existent ou non pour lutter contre ce phénomène ; si tel était le cas, la le narcotrafic s’épanouit partout où l’État central déserte. Par endroits, il a même pris le relais de l’État. Je vous invite à aller voir ce qui se passe actuellement en Argentine, où la dépense publique a véritablement été coupée à la tronçonneuse, ce qui semble en faire rêver plus d’un scolaires dans ce que l’on appelle les « villes misère » ? Ce sont les narcotrafiquants : ils ne se glissent pas seulement dans chaque faille juridique, mais également dans chaque faille sociale, créant une dépendance et une soumission économiques des populations avec lesquelles ils vivent et dont ils font partie. Les narcotrafiquants deviennent, de fait, pour les adolescents, le seul modèle de succès auquel ils aspirent, simplement parce qu’il est le seul auquel ils peuvent prétendre. Nous pourrons difficilement nous donner les moyens de « sortir du piège du narcotrafic » sans renforcer l’ensemble des services publics permettant d’éviter qu’un gamin ne tombe dedans. C’est parce que ce texte prévoit plus d’État dans un domaine qui en a cruellement besoin que le groupe RDSE votera pour son adoption. Il nous permet de commencer à rattraper un retard certain ; il devra s’accompagner des moyens humains indispensables pour mener à bien cette mission.

300 millions de consommateurs, la majorité des usagers consomment du cannabis, 60 millions des opioïdes, 30 millions des amphétamines, etc. pour un chiffre d’affaires consolidé de 250 milliards de dollars. Dans ce contexte, la situation en Syrie, terre du Captagon,

notre collègue Pascal Martin, visant à permettre le bannissement des ports français des navires impliqués dans le trafic de stupéfiants et, par extension, des compagnies qui les utilisent. Moins de drogue au Havre, c’est moins de drogue dans l’Orne, monsieur le président ! Je souhaite

À la longue liste des failles qui existent, il faut ajouter : les ports francs, les paradis fiscaux et nos amis des monarchies du Golfe, qui ont leur propre modèle économique.

Jérémy Bacchi, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste

Je pense bien sûr aux dockers, aux salariés des ports, aux douaniers, aux agents pénitentiaires, aux avocats, aux magistrats, aux policiers, aux gendarmes et à tant d’autres. C’est notre devoir que de les protéger face aux risques qu’ils affrontent chaque jour. Nous devons prendre garde à garantir leur sécurité, tout en proportionnant les contrôles dont ils font l’objet. Nous ne pouvons pas les présumer complices, et encore moins coupables ; au contraire, il nous faut tout mettre en œuvre pour les préserver contre les risques de corruption ou les menaces liés au trafic de drogue. Je regrette d’ailleurs ici que les amendements que nous avions déposés en ce sens n’aient pas été retenus. J’espère que le travail législatif qui suit son cours réparera ce manquement. Je souhaite aussi rendre hommage aux travailleurs de l’aide sociale à l’enfance

les poussons dans les bras des narcotrafiquants et des proxénètes. Il devient urgent de soutenir financièrement nos départements pour mieux protéger ces enfants. Si nous ne renforçons pas le secteur de la protection de l’enfance, nos efforts seront vains. Je souhaite enfin rendre hommage aux habitantes et aux habitants des quartiers, des villes et des villages touchés par ce fléau que nous combattons ici. nous combattons ici. Il nous faudra prendre garde, en cherchant à les protéger, à ne pas les enfermer dans un quotidien uniquement sécuritaire et marginalisant. J’ai grandi dans les quartiers nord de Marseille et je sais que nous ne pouvons pas être réduits à cela : nos quartiers sont beaux et peuvent nous rendre fiers.

Partout sur le territoire national, la présence de l’État doit être renforcée, notamment au travers du développement des services publics. En tant que communiste, je sais que la lutte contre les mafias est une question de classe. Les premières victimes des réseaux mafieux sont les populations les plus fragilisées, les plus vulnérables et les plus précaires. Lorsque l’État les abandonne, les trafiquants se montrent bien présents, gangrenant notre pays et profitant des failles ouvertes. Et partout où l’État recule, les mafias progressent.

Quand la France dépense 77 euros par an et par habitant pour sa justice, l’Espagne dépense 96 euros, l’Italie 100 euros et l’Allemagne 136 euros. Concrètement, la France ne compte que 11,3 magistrats professionnels pour 100 000 habitants, contre 24,17 en Allemagne, soit plus du double.

Enfin, même si la question de la prévention et des usagers de drogue n’est pas l’objet de cette proposition de loi, il nous faudra mener une véritable campagne de santé publique pour soigner ces personnes de plus en plus nombreuses et de moins en moins accompagnées.

mais étendues à l’ensemble de la criminalité organisée. Notre groupe salue cette vision à la juste échelle de ces nouvelles mafias, auxquelles il est nécessaire d’accorder une attention particulière. Nous alertons cependant sur la dérive possible vers une centralisation excessive, car nous devons être conscients que ces criminalités se retrouvent sur l’ensemble du territoire, en zone urbaine comme en zone rurale, de Marseille à Morlaix en passant par la Corrèze et la région parisienne.

Pour être véritablement dissuasive, toute sanction pénale doit pouvoir s’accompagner de la privation des délinquants des profits qu’ils ont pu tirer de l’infraction. » Taper au portefeuille, faire en sorte que le crime ne paie pas

de la focalisation sur le haut du spectre, nous nous félicitons de la refonte et de la sécurisation du statut de ceux que l’on nomme communément les repentis et de l’adoption de l’un de nos amendements tendant à mieux les protéger en sanctionnant ceux qui révèlent des informations sur les repentis et leurs proches.

Rien sur les mesures d’information permettant d’éviter l’entrée dans la consommation. Rien sur les parcours de soins, sur la prise en charge des addictions, sur l’intérêt de légaliser ou de dépénaliser certains usages. Aucune mesure de politique de santé publique.

ailleurs, quelques points de ce texte sont très problématiques. Nous sommes notamment stupéfaits d’avoir vu réapparaître les mesures d’activation à distance des appareils électroniques dans le but de capter les conversations.

dans la mesure où elle permet l’enregistrement […] concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers. » Nous restons également convaincus que les mesures dérogatoires permettant l’allongement des délais de détention provisoire ou de garde à vue sont disproportionnées. nous déplorons l’adoption de l’article 24, absolument absent des conclusions et préconisations de notre commission d’enquête, qui vise à mettre en place des mesures à la fois inopérantes et inefficaces. Nous espérons que la navette parlementaire permettra de revenir sur ces articles au mieux inutiles, voire dangereux pour l’équilibre entre la lutte légitime contre le narcotrafic et la garantie, tout aussi légitime, des droits de la défense et des libertés individuelles.

Monsieur le président, messieurs les ministres d’État, mes chers collègues, ce texte est né de Marseille, j’irai par conséquent « droit au but » : notre groupe votera pour cette proposition de loi.

À Paris, Rennes, Nantes, Saint Ouen, Clermont Ferrand, Fort de France, Montpellier, Nancy, Vesoul, Lille, dans les centres des métropoles, dans les villes moyennes ou dans les campagnes, nos élus locaux font face à la violence, aux morts et à la déstabilisation opérée par le trafic de drogue. Un fléau dont on a trop longtemps cru qu’il était réservé à certains territoires. Le terrorisme fracasse la société, nous savons désormais que le narcotrafic la ronge. Il est question de victimes humaines, de territoires sous emprise et d’une menace pour la démocratie. Je veux remercier Marie Arlette Carlotti pour avoir, la première, avec ses collègues Jérémy Bacchi et Guy Benarroche, milité pour que le Sénat s’attaque avec pugnacité à ce phénomène. Valérie Boyer et Stéphane Le Rudulier ont ensuite obtenu la création de la commission d’enquête Grâce à ces sénateurs de gauche et de droite investis dans la commission d’enquête, qui a rendu ses conclusions en mai dernier, une volonté s’est exprimée de faire front ensemble, partout, face au piège qui nous guette. Il nous fallait ensuite traduire dans la loi ces préconisations. C’est une grande fierté d’avoir pu assumer la copaternité, avec mon collègue Étienne Blanc, de cette proposition de loi. Nous n’avons ni le même parcours ni les mêmes orientations politiques, mais ce travail transpartisan nous a semblé naturel et indispensable. Mieux, il incarne pour nous le meilleur de ce que peut apporter le travail parlementaire. Nous avons partagé tout au long de ces travaux la conviction sincère qu’il fallait avancer vite et fort. Cela nous a conduits parfois à empiéter sur le pré carré de l’exécutif, dans une démarche d’autant plus inhabituelle qu’elle concerne le cœur des missions régaliennes. Ce texte Ce texte comprend deux volets : d’abord, une organisation repensée de la lutte contre le narcotrafic autour de deux chefs de file, l’un judiciaire, l’autre dans l’investigation ; ensuite, une exceptionnelle boîte à outils, qui donne à notre première ligne des moyens juridiques et techniques nouveaux. Corruption, blanchiment, procédure pénale, renseignement, techniques d’enquêtes… Que ce soit la mise en place du procès verbal distinct, la réforme du statut des repentis, l’injonction pour richesse inexpliquée, l’infiltration civile ou encore la nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle, les nouveaux outils ne manquent pas. Ils étaient réclamés massivement par les magistrats, les policiers, les gendarmes, les douaniers, tous les spécialistes que nous avons auditionnés pendant ces longs mois de travaux. Charge maintenant à l’Assemblée nationale de consolider leur inscription dans la loi. Notre groupe a pris toute sa part dans cette construction. Je veux évoquer ici : un meilleur maillage contre le blanchiment, grâce à Hussein Bourgi ; une meilleure protection de l’identité des professionnels de la justice en cas de menace, ou encore la protection des informateurs, grâce à Marie Pierre de La Gontrie ; une lutte renforcée contre la corruption, grâce à Marie Arlette Carlotti ; une meilleure prise en compte des spécificités ultramarines, grâce à Catherine Conconne Conconne et Victorin Lurel ; l’amélioration de la lutte contre le trafic en prison, grâce à Laurence Harribey ; ou encore la lutte contre l’utilisation massive de cartes SIM prépayées par les trafiquants, grâce à Corinne Narassiguin. S’agissant de lutte contre le crime, les sénatrices et sénateurs socialistes ont toujours recherché le nécessaire équilibre entre sécurité et liberté. Comme lorsque nous avons affronté la question du terrorisme, il a fallu procéder à des arbitrages difficiles. L’alpiniste que je suis connaît la difficulté des parcours d’arête ; arpenter la ligne de crête est toujours périlleux. Dans ce tableau globalement positif, il me faut ici exprimer quelques frustrations, quelques agacements et une franche opposition. Nos réserves se sont concentrées sur l’article 16, relatif au procès verbal distinct, ou encore sur le régime des nullités de l’article 20. Nous estimions que le travail réalisé par la commission des lois et sa présidente permettait d’atteindre un équilibre satisfaisant, par une rédaction clarifiée et sécurisée. D’une manière générale, trop d’amendements gouvernementaux sont arrivés bien trop tard et leur portée aurait mérité un débat plus approfondi. Nous avons cependant confiance en la navette parlementaire pour qu’un équilibre encore meilleur vienne concrétiser l’engagement sur ce texte

Un dispositif à ce point intrusif mériterait une étude d’impact approfondie, une préparation minutieuse et un débat parlementaire nourri. Très bien ! Nous n’avons rien eu de tout cela. Cet amendement aurait dû être défendu par le Gouvernement dans un texte consacré au renseignement. Vous connaissez l’attachement de la gauche au service public. Il faut protéger nos concitoyens de la gangrène du narcotrafic et aider nos maires démunis. Mais il ne peut y avoir d’État protecteur avec des forces sous dotées, une justice embolisée et des prisons cocottes minute. Vous l’aurez compris : nous demandons des moyens. Le parquet national anti criminalité organisée et le nouvel état major annoncé par les ministres Retailleau et Darmanin, constituent des incarnations et des outils de coordination bienvenus et indispensables. Mais ils ne seront fonctionnels que s’ils sont dotés des moyens suffisants en termes humains et d’équipements. La menace que fait peser le narcotrafic sur les intérêts fondamentaux de la Nation le justifie. L’investissement sans faille des enquêteurs et magistrats, partout sur le terrain, nous engage. Il appelle de notre part un soutien entier, y compris sur le plan budgétaire.

afin de conserver un consensus transpartisan le plus large possible. Comme l’a rappelé Audrey Linkenheld, notre groupe considère qu’il faut avancer sur deux jambes. La jambe répressive, nous l’assumons sans fard ; celle de la prévention et du soin, nous l’appelons de nos vœux. La drogue concerne un nombre important de criminels et un nombre encore plus important de victimes. nous faut combattre les criminels de toutes nos forces, il faut aussi soigner et accompagner les consommateurs, qui peuvent être dépendants et malades. C’est pour nous une priorité et nous formulerons bientôt des propositions en ce sens. Pour l’heure, les socialistes sont à leur place en votant le soutien à tous ceux qui combattent en notre nom, au quotidien, la criminalité organisée.

Monsieur le président, messieurs les ministres d’État, mes chers collègues, l’examen de la proposition de loi transpartisane sur le sujet majeur que constitue notre combat contre le narcotrafic me fournit l’occasion de saluer le travail de nos collègues Étienne Blanc et Jérôme Durain ainsi que celui des membres de la commission d’enquête.

Je salue l’esprit de responsabilité qui a dans l’ensemble animé nos débats sur un sujet depuis longtemps dénoncé par le Rassemblement national. La proposition de loi devra s’appliquer et se traduire par des résultats concrets. Nous avons beaucoup d’espoir dans le renforcement de l’Office anti stupéfiants, composé de quatre ministères régaliens – Beauvau, Bercy, place Vendôme, les armées. Nous souhaitons que leurs services sachent travailler et coopérer. Avec ce Avec ce texte, nous frapperons enfin les narcotrafiquants au portefeuille en systématisant les enquêtes patrimoniales et en créant une nouvelle procédure d’injonction pour richesse inexpliquée.

Il faut en effet parler de fléau quand pas moins de 80 % des règlements de compte par armes à feu dans notre pays sont le fait du narcotrafic. Désormais, plus aucun territoire n’est désormais épargné. Le Premier

messieurs les ministres d’État, mes chers collègues,

Si vous disposez d’une délégation de vote, le nom du sénateur pour lequel vous devez voter s’affiche automatiquement sur le terminal en dessous de votre nom. Vous pouvez alors voter pour vous et pour le délégant en sélectionnant le nom correspondant puis en choisissant une position de vote.

l’ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti stupéfiants,

je vais donner la parole à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

l’absence de distinction et d’identification de la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un marché global conduirait à priver l’architecte de toute marge de manœuvre et d’expertise indépendante vis à vis de l’opérateur économique.

de sécuriser l’expertise des architectes mahorais. Ils sont une trentaine à être inscrits à l’ordre, dont vingt sont formés à la gestion de crise en collaboration avec la fondation Architectes de l’urgence.

contre

Dans un territoire où le taux de chômage atteint 37 % et où la jeunesse désespère de trouver du travail, il serait inconcevable que les chantiers profitent uniquement aux grands groupes de BTP de l’Hexagone. Mayotte dispose de toutes ses forces vives pour se reconstruire elle même. Nous devons lui proposer de l’ingénierie juridique et technique, tenir à sa disposition les moyens financiers nécessaires et permettre les transferts de compétences.

n° 119 rectifié. Pour préserver les acteurs économiques locaux, particulièrement les entreprises artisanales mahoraises du bâtiment, cet amendement vise à limiter la sous traitance à deux rangs L’objectif est de lutter contre la sous traitance en cascade, qui fait courir un risque sur la qualité soit des travaux réalisés soit des matériaux utilisés, en raison souvent d’une extrême tension sur les prix d’un rang à l’autre. Les défauts de qualité affectent la conformité des ouvrages, donc les services rendus aux particuliers. Plus globalement, ils risquent de nuire à toute reconstruction durable et harmonieuse de Mayotte. la sous traitance en cascade grève la valeur ajoutée d’un rang à l’autre et entraîne une paupérisation de l’ensemble de la chaîne de valeur, ce qui fragilise fortement les entreprises artisanales du bâtiment.

Pour faire face aux défis qui s’annoncent, pouvoir compter sur la connaissance du territoire, sur le savoir faire des artisans et sur leur mobilisation rapide grâce à leur proximité, y compris pour assurer le suivi des travaux, À l’inverse, si des entreprises extérieures devaient être privilégiées pour répondre aux appels d’offres à venir, certains artisans locaux ne s’en relèveraient pas, alors que plusieurs d’entre eux connaissent déjà de grandes difficultés.

actuelle permettrait aux entreprises capables de répondre à des marchés supérieurs à 300 000 euros de s’exonérer d’un plan de sous traitance. De fait, il est plus simple pour elles de déléguer les missions du marché une fois que celui ci leur a été attribué. Cette disposition ne se justifie pas,

d’obliger les petites entreprises à se doter d’un plan de sous traitance, ce qui alourdirait leur charge administrative de manière excessive, et, d’autre part, de ralentir

besoin que Paris fasse enfin confiance à Mayotte.

massivement. Ensuite, la limitation de la sous traitance risque de bloquer complètement l’accès à la commande publique des artisans et travailleurs indépendants, qui n’ont pas la capacité d’agir en tant qu’entreprise principale. N’oublions pas que l’article 11, que nous avons examiné hier, a offert la possibilité de négocier de gré à gré dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone, si la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros.

Je tiens à souligner que le tissu économique local est fragile. Il a évidemment besoin de soutien. Faisons donc attention aux mesures dont les principes sont louables – je les partage –, mais qui peuvent être en décalage avec la réalité économique du terrain.

aller dans ce sens. C’est l’objet des amendements qui vous sont proposés. L’État, les organisations patronales et l’ensemble des corps intermédiaires doivent pouvoir accompagner la montée en compétences des TPE PME mahoraises pour les aider à se relever de façon robuste après le cyclone Chido.

et solidaire (ESS) est bien présent à Mayotte et se dit prêt à contribuer à la reconstruction du territoire. Dès lors que le code de la commande publique n’y fait pas obstacle, le présent amendement vise à garantir une intégration de l’ESS au sein de cette réserve. L’ESS représente à Mayotte 14 % des entreprises, soit 281 structures, et 23 % de l’emploi privé. À Mayotte, les associations de l’ESS sont actives, créatives et productives. Outre le fait qu’elles puissent aisément répondre aux appels d’offres en matière de nettoyage, par exemple, elles pourront, grâce à leur expertise, identifier ce qui est susceptible d’être valorisé afin de donner une nouvelle vie aux matériaux récupérables.

Vous avez raison, madame la sénatrice, de souligner l’importance du tissu de l’économie sociale et solidaire mahoraise. Ce secteur, dont vous avez rappelé les chiffres, aura un rôle important à jouer dans la reconstruction de Mayotte.

Les apprentis peinent à trouver des structures d’accueil pour assurer leur formation pratique. La réserve de 30 % pour ces entreprises vise à garantir un esprit de solidarité et de partage de la ressource. amendement tend à les impliquer à leur tour dans cet effort de transmission et de formation, indispensable pour l’avenir de la jeunesse mahoraise, qui bénéficie d’une occasion d’être formée dès la rentrée prochaine. Il y a urgence à investir dans l’acquisition de compétences par la jeunesse, dans le secteur du BTP.

un avis défavorable

de cet amendement. En effet, le dispositif proposé risque de bloquer l’exécution des travaux de reconstruction de Mayotte et de ralentir la passation des marchés publics. En effet, dans le cas où aucune entreprise n’utiliserait des matériaux biosourcés ou bas carbone, il ne serait pas possible d’exécuter puisque le titulaire du marché public ne pourrait sous traiter une partie du marché à des entreprises respectant ces critères. De plus, en l’état, la rédaction de l’amendement n’a pas l’effet annoncé dans l’objet : il se contente de prévoir une obligation de sous traitance à des PME ou à des artisans

proposons un dispositif permettant de réduire cette dépendance et de faire en sorte qu’une partie des matériaux soit de provenance régionale. Cela permettrait également de réduire l’impact carbone lié à l’importation de matériaux de construction.

Les forêts de Madagascar ou du Mozambique pourraient fournir le bois nécessaire à la reconstruction. Cela ne signifie pas que nous voulons réduire les exigences environnementales et sociales. En tant qu’écologistes, nous sommes très vigilants sur cette question. Nous connaissons la situation des défenseurs de la biodiversité dans certains États voisins,

de production. Les territoires ultramarins peuvent devenir les ambassadeurs du droit de l’environnement européen, en engageant des dialogues avec des États voisins. Ce dispositif temporaire pourrait permettre d’évaluer si l’intensification des relations commerciales

Evelyne Corbière Naminzo. L’article 13 a été supprimé en commission au motif, notamment, qu’il fallait respecter le principe de libre recours à la sous traitance. Ce libre recours mène pourtant à des dérives,

L’urgence que rencontre Mayotte ne doit pas être une aubaine pour les multinationales du BTP – nous en savons quelque chose, nous autres Ultramarins ! Au contraire, il importe de s’appuyer sur les entreprises mahoraises pour ne pas aggraver la crise économique économique déjà présente avant le cyclone et qui se trouve aujourd’hui renforcée. C’est en ce sens que nous proposons de rétablir l’article 13 en limitant la sous traitance à deux rangs afin d’éviter un éloignement trop important entre les entreprises lauréates donneuses d’ordre et les entreprises exécutantes.

ans. Il paraît raisonnable de soutenir le tissu économique local de façon générale et pérenne si nous voulons permettre à Mayotte d’avoir le développement qu’elle mérite.

l’article 14 tend à prévoir que les dérogations aux règles de la commande publique s’appliqueront aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur du présent texte. Cette précision vise un objectif de sécurité juridique pour éviter que les règles ne changent subitement pour les marchés

Ramia. Afin de veiller à la bonne utilisation des deniers publics, le présent amendement tend à prévoir que les associations et fondations reconnues d’utilité publique ayant bénéficié de subventions de de la part des collectivités territoriales ou de leurs groupements devront établir un rapport d’activité, au plus tard le 1 mars 2026. Ce rapport présentera les actions financées grâce aux subventions versées par les collectivités territoriales et précisera le nombre de bénéficiaires de chaque action, ainsi que la nature de la prestation fournie. Ce rapport d’activité devra ensuite être rendu public, dans un objectif de transparence.

Cet amendement vise donc à prolonger jusqu’à la fin de l’année 2025 le dispositif fiscal exceptionnel, qui encourage la générosité des Français en faveur de Mayotte en portant la réduction d’impôt sur les dons de 66 % à 75 %. Cette prolongation répond à un double impératif : un besoin opérationnel, pour garantir des ressources suffisantes pour la reconstruction

délibérément courte pour renforcer son caractère incitatif et engendrer un surcroît de dons. En outre, passé cette date, les dons bénéficient toujours du taux majoré pour les actions de fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté d’amélioration des conditions de logement et de fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté – c’est le dispositif dit Coluche de droit commun –, la seule différence étant que ces dons ne seront plus exclus du calcul total des dons effectués par un particulier à des associations pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable, qui s’applique à cette réduction d’impôt.

Dès le lendemain du passage de Chido, les associations étaient à pied d’œuvre pour apporter de l’aide à la population mahoraise. À juste titre, l’article 16 de ce projet de loi tend à augmenter la réduction d’impôt accordée aux dons à ces associations pour soutenir le travail sur le terrain. Ces trois amendements visent à étendre le périmètre des associations éligibles à ces réductions d’impôt en permettant d’abord de soutenir les associations qui œuvrent à l’amélioration de l’habitat des personnes, y compris celles qui vivent dans des habitats informels.

convient de soutenir les associations qui œuvrent dans deux champs aujourd’hui ignorés par ce projet de loi : les associations qui participent au reboisement de l’île et celles qui travaillent à la conservation du patrimoine culturel mahorais.

rectifié, la réduction d’impôt majorée prévue à cet article vise à encourager les dons des particuliers pour la mise en œuvre de mesures d’urgence de soutien aux populations éprouvées par le passage du cyclone. Les dons aux associations qui œuvrent au reboisement, au maintien ou au développement de la biodiversité ouvrent déjà droit, dans les conditions de droit commun, à une réduction d’impôt de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

pour tous les sujets, aussi importants soient ils. Les dons aux œuvres et organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel ouvrent déjà droit, dans les conditions de droit commun, à une réduction de 66 %, dans de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. C’est le cas, par exemple, des dons à la Fondation du patrimoine, qui mène plusieurs projets à Mayotte, ou à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées intervenant dans le domaine de la protection du patrimoine.

amendement vise à encourager les dons des particuliers destinés à la reconstruction de Mayotte.

encore, les travaux n’ayant pas vraiment démarré. Au demeurant, si nous pouvons chiffrer ces dégâts à plus de 1 milliard d’euros, combien d’argent faudra t il pour que la reconstruction soit ambitieuse ? Celle que nous appelons de nos vœux doit permettre de mieux faire face aux prochaines catastrophes qui risquent de se produire, compte tenu du dérèglement climatique et de ses effets destructeurs. Aussi, pour favoriser les dons aux associations et aux fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte, à la suite du Cyclone Chido, fournissent déjà gratuitement des repas et des soins aux personnes en difficulté et contribuent à favoriser leur relogement,

à ces trois amendements, pour trois raisons. Premièrement, les dispositions en vigueur ouvrent déjà droit à réduction d’impôt pour les dons des entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent à titre principal à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins ou de matériel nécessaire pour vivre décemment, ce qui permet de couvrir la majeure partie des besoins visés. Deuxièmement, je que cette mesure, contrairement à celle qui concerne les particuliers, n’a pas été annoncée dès le mois de décembre 2024. Or mettre en place une telle mesure fiscale incitative à titre rétroactif est pour le moins contestable.

d’engager rapidement les travaux. Nous savons, puisque nos amendements ont été rejetés, que beaucoup de cet argent ira droit aux majors du BTP.

C’est fort dommage

Quelques jours après Chido, le représentant de l’État, dans une intervention publique, a évoqué sa crainte de centaines, voire de milliers de victimes. De surcroît, il a évoqué notre rite musulman d’un enterrement des corps sous vingt quatre heures, sous entendant, fort justement d’ailleurs, que des victimes auraient pu échapper à la procédure normale d’une déclaration après un décès.

Je n’ai pas obtenu de réponse précise à ma demande, sinon un tableau global des bilans, des « aller vers », mais rien sur le résultat des recherches des disparus. Vous comprendrez que ce culte du secret développe un sentiment de suspicion à l’égard de l’État. Je sais que vous n’êtes pas indifférent à Mayotte, que vous connaissez notre archipel.

pourra, à mon sens, être fait dans un second temps : avis défavorable.

repose sur un lien avec les communes et une prise de pouls régulière de chacune d’entre elles. J’ai encore pu le constater sur place, avec les maires. Ces revues de territoire permettent également de rendre compte de l’action de l’État. Je pense également aux conférences de sécurité, organisées régulièrement pour rendre compte de l’action de l’État en matière de lutte contre l’insécurité, contre l’économie souterraine, contre l’immigration clandestine, auxquelles les maires sont conviés. Ces deux exemples parmi d’autres illustrent que l’État rend compte de son action. Pour refonder Mayotte, il faut de la cohésion et de l’unité. Si la défiance existait avant Chido – non pas à l’égard du préfet, mais entre les Mahorais, les élus et l’État hexagonal

Il faut rappeler que, par peur d’être piégés, contrôlés, expulsés, de nombreux habitants en situation irrégulière ne se sont pas rendus dans les abris. L’État, aux yeux d’un grand nombre de personnes sans papiers, n’a pas été protecteur.

le préfet, lui, a failli… être écrasé par l’effondrement du toit du centre de crise au cœur du passage du cyclone ! Mesdames, messieurs les sénateurs, remettons certaines déclarations dans leur contexte,

l’appui du Gouvernement, tend à lever les gages qui ont été ajoutés à cette occasion à l’article 17.

ministre du plan Mayotte debout. Le montant du prêt ne pourra pas excéder 50 000 euros par logement et sa durée de remboursement pourra être de trente ans, avec un différé de remboursement de cinq ans maximum pour les publics les plus fragiles. de parfaire le dispositif et de soutenir les Mahorais dans la reconstruction de leur logement, le prêt sera garanti par l’État. Enfin, ce dispositif rétroactif sera limité dans le temps et s’appliquera aux prêts demandés jusqu’au 31 décembre 2027.

dans les mêmes conditions que pour les employeurs et artisans, commerçants et non salariés agricoles et maritimes, y compris pour ce qui concerne les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité décès. La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les sections professionnelles des professions libérales se sont déjà montrées favorables à un tel dispositif. de décaler les dates d’octroi des plans, afin que les caisses de sécurité sociale aient le temps de rassembler les informations sur la situation des cotisants, notamment en ce qui concerne les travailleurs indépendants, dont la dette contractée en 2025 ne pourra être connue

Cette faculté, qui tire les leçons des expériences de l’ouragan Irma et de la crise sanitaire, permettra de s’adapter au plus près à la situation financière des entreprises locales.

L’Assemblée nationale avait ajouté à l’article 18 des dispositions introduites à la suite du passage du cyclone Irma à Saint Barthélemy. Elles prévoyaient la possibilité de conclure des plans d’apurement de cotisations entre les redevables et les organismes de recouvrement.

Dans le texte de la commission, la suspension de droit a pourtant été ramenée à son terme initial, soit au 31 mars 2025. Cette nouvelle échéance envoie un message délétère aux acteurs économiques, qu’elle abandonne à leur résilience. Elle complexifie et fragilise grandement la conclusion de plans d’apurement des dettes, qui permettraient d’assainir de manière pérenne la situation des entreprises locales. Aussi, le présent amendement tend à étendre la période relative à la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales jusqu’au 31 décembre 2025, avec possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu’au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie. Ce second point est essentiel pour sécuriser les entreprises et les emplois mahorais.

travailleurs indépendants et microentrepreneurs mahorais, afin de leur octroyer un sursis nécessaire pour faire face aux dépenses induites par le cyclone Chido. La commission a modifié cet article afin de revenir aux échéances initialement prévues dans ce texte

Le secteur bancaire fonctionne normalement et les collectivités vont pouvoir passer des commandes importantes pour la reconstruction des structures publiques. Dans ces conditions, il ne me semble pas raisonnable de suspendre le recouvrement des cotisations pendant presque deux ans. Je rappelle également que les dispositions de l’article 18 protègent déjà largement les acteurs économiques vulnérables, en permettant l’abandon pur et simple des cotisations dues au titre des exercices 2024 et 2025 pour les travailleurs indépendants

Les petites entreprises locales sont confrontées à un manque de financement et à des difficultés d’accès au marché extérieur, ce qui limite leur capacité à se développer et à créer des emplois durables. Or le projet de loi d’urgence que nous examinons ne les favorisera Les travailleurs indépendants dans les secteurs agricole et maritime font face à une situation économique fragile et à des difficultés structurelles. Ainsi, la majorité des exploitants agricoles sont des producteurs de petite échelle, qui peinent à diversifier leurs cultures.

Cet amendement a été très bien défendu à l’instant. Ce dispositif exceptionnel de suspension de paiement va dans le bon sens, mais souffre de conditions d’application peu adaptées à la gravité de la crise provoquée localement par le cyclone Chido. Par ailleurs, les intempéries se poursuivent. Dans ce contexte, la suspension des cotisations pour l’ensemble des entreprises jusqu’au

Je le répète, si les secteurs sont inégalement touchés, certains indiquent déjà qu’ils pourront reprendre rapidement leur activité. Certains commerces ont été épargnés par le cyclone et voient leur chiffre d’affaires augmenter. En raison de l’afflux de clientèle, le BTP sera quant à lui fortement mobilisé pour reconstruire ce qui a été détruit. La mesure de suspension actuellement prévue me semble donc suffisante, car elle protège les plus vulnérables et leur offre déjà la possibilité de bénéficier d’un abandon de créances de cotisations, à la condition de démontrer l’impact durable du cyclone sur leur activité. Enfin,

telles qu’une exonération complète. Ce type de dispositif avait déjà été mis en place durant la crise sanitaire liée à la covid 19 pour les secteurs fortement touchés par les confinements, comme le tourisme et la restauration. Compte tenu de la quasi paralysie

Mme Raymonde Poncet Monge. Depuis plusieurs mois, on observe la même scène à Mamoudzou, la capitale de l’île : le jour à peine levé, des dizaines d’habitants se précipitent pour faire la queue devant des conteneurs. Dans ces caissons métalliques se trouve une ressource vitale qui se fait de plus en plus rare : des packs d’eau potable. Avoir de l’eau potable à Mayotte est vraiment compliqué. On essaie de trouver des packs d’eau dans les supermarchés, mais il n’y en a pas toujours et ça coûte cher. » Ces mots d’un

Aujourd’hui, l’accès à l’eau et à des produits de première nécessité est restreint dans l’archipel. Les distributions d’eau sont insuffisantes. Cet amendement vise à garantir l’accès à l’eau et aux produits de première nécessité durant ces semaines d’urgence,

du plan Eau de Mayotte. Cet ingénieur en chef, spécialisé dans les métiers de l’eau, aura comme objectif le rétablissement d’un service d’eau potable de qualité dans le département. Le général Facon, qui était encore sur place aujourd’hui,

Mme Raymonde Poncet Monge. L’objet de cet amendement est de rétablir l’article 27. Alors qu’une convergence sociale a été annoncée par le Gouvernement, nous demandons l’instauration d’un calendrier d’alignement des prestations sociales sur celles de l’Hexagone.

De même, selon l’Insee, le système redistributif public ne réduit que très marginalement la pauvreté à Mayotte. Les prestations sociales ne font baisser le taux de

Les inégalités entre l’Hexagone et Mayotte concernent non seulement les conditions de vie ou le pouvoir d’achat, mais également les prestations sociales, dont l’objet est pourtant de réduire ces inégalités. Nous savons que la catastrophe

Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, d’une part, sur le bilan de la prolongation des droits versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d’autre part, sur la nécessité de suspendre à Mayotte les dernières réformes de l’assurance chômage. L’avis est défavorable, car cet amendement vise à rétablir un article supprimé en commission. de la position constante de la commission sur les demandes de rapport, les réformes récentes de l’indemnisation du chômage se trouvent de fait suspendues le temps de la prolongation automatique de l’allocation de retour à l’emploi. Si des mesures s’avéraient nécessaires pour le retour au régime de droit commun, il incomberait alors aux partenaires sociaux de déterminer les ajustements utiles aux règles d’assurance chômage. Ce rapport n’est donc pas souhaitable.

de la gestion des déchets. Nous suivrons également de près la replantation de la forêt mahoraise et le soutien apporté à l’agriculture de Mayotte, durement touchée. Nous espérons que l’article 13 AA, qui permet aux TPE de répondre aux marchés publics, sera maintenu. Il protège la liberté d’entreprendre, mais, surtout, il garantit à ces entreprises le droit d’exister. Nous le savons, le tissu d’outre mer est fragile et souvent à la merci des monopoles et des. Pour nous, il faut permettre aux forces vives mahoraises de piloter la reconstruction. Nous regrettons que les débats soient encore trop orientés sur la problématique migratoire, comme si l’on cherchait à rejeter la responsabilité de la gravité des dégâts causés par Chido sur les personnes en situation irrégulière. C’est oublier que Mayotte est le département de l’injustice sociale et des promesses non tenues, avec des droits sociaux bafoués, que ce soit pour les allocations familiales, pour les personnes porteuses de handicap ou le RSA,

ne puissent pas faire autrement que de s’abriter dans des bidonvilles, en achetant des tôles grâce à leur carte d’identité française… Nous voulions tous que ce texte remette Mayotte debout, mais, déjà, les fondations de cette reconstruction valident une société qui discrimine, que ce soit entre citoyens français – ceux de Mayotte et ceux d’ailleurs –, entre Mahorais – les plus précaires et les autres

Les propos d’Emmanuel Macron après le passage du cyclone résonnent encore tant ils relèvent inconsciemment d’un regard colonial brutal. Il aurait fallu que les Mahoraises et les Mahorais, habitants d’une ancienne colonie départementalisée en 2011, soient contents d’être Français… Mais est on sûr que la dette est de leur côté ? Malgré une République prétendument égalitaire, Mayotte n’est pas le territoire de l’égalité des droits. Comme pour M. Macron, la

Il nous faut urgemment prendre en compte ce que le chercheur Malcolm Ferdinand appelle une double fracture environnementale et coloniale qui résonne encore, les inégalités se perpétuant entre l’Hexagone et les territoires ultramarins. Bernard Kalaora, socioanthropologue, explique de son côté que les Mahorais, exclus de l’élaboration du projet de protection de l’écosystème marin du parc naturel de Mayotte – en tant qu’écologistes, nous sommes très attachés à ce parc –, perçoivent cette conservation comme une « colonisation bleue où la priorité est donnée à la nature administrée par l’État français au détriment des habitants. Oui, ce qui est fait sans les Mahoraises et les Mahorais se fait contre eux. Pour le chercheur, la situation actuelle peut être qualifiée d’« hypercriticité », « un état où les tensions sociales, politiques et environnementales atteignent un point de rupture, où chaque élément peut précipiter

et nous comptons sur le futur projet de loi qui est annoncé pour travailler sur les points fondamentaux que nous n’avons pas pu aborder ici à cause d’une application très stricte de l’article 45.

à l’issue de l’examen de ce texte, pouvons nous dire en toute honnêteté que nous avons trouvé toutes les solutions concrètes pour un archipel ravagé ? Que nous avons répondu aux besoins d’une population soumise à toutes les vulnérabilités ? Que nous avons pris en compte la réalité inacceptable de ces enfants qui ne sont scolarisés que lorsqu’ils le peuvent, et non lorsqu’ils le doivent ? Que nous avons soutenu les forces vives mahoraises, les entreprises, les artisans, qui eux aussi sont capables de reconstruire leur territoire Que nous avons anticipé les prochaines fureurs climatiques, préservé une faune et une flore d’une richesse incroyable ? Que nous avons garanti un accès à l’eau aux 28 % de logements qui en étaient déjà privés ? Que nous avons traité avec égalité toutes les victimes de ce cyclone ? Que le montant alloué à cette reconstruction est suffisant

Mais en réalité, cela ne change pas la réponse à toutes ces questions. Alors oui, nous concernant, nous allons voter ce texte et vous donner les moyens de répondre en partie à l’urgence. Non pas parce que nous partageons votre méthode : nous refusons de sanctionner les sans papiers, qui sont des victimes de ce cyclone tout autant que les autres. Nous le voterons, parce que nous refusons de laisser les Mahoraises et les Mahorais s’enfoncer encore plus dans la détresse.

l’éducation, l’eau – et j’en passe… Mes chers collègues, Mayotte ne mérite pas une vision hors sol pour se reconstruire. Les délégations successives en visite sur place ne peuvent que constater, sur le terrain, ce à quoi font face les Mahorais au quotidien : Mayotte arrive à une situation de saturation ; sa population, qui est accueillante, est à bout de souffle.

à la réalité du territoire mahorais et associer le plus possible les élus. Je tiens à rendre un hommage tout particulier à nos deux collègues mahorais,

aucune raison de masquer la vérité, en tout cas celle qui est connue aujourd’hui. Je veux aussi vous remercier, parce que vous vous êtes déjà rendu plusieurs fois à Mayotte et que vous continuerez à vous y rendre. Le Sénat restera bien évidemment mobilisé pour les Mahoraises et les Mahorais

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, nous y sommes enfin Plus d’un an après avoir été promis à nos agriculteurs, plus de onze mois après son dépôt en conseil des ministres, près de neuf mois après son vote en première lecture à l’Assemblée nationale, le projet de loi d’orientation agricole voit enfin s’engager son Il s’agit maintenant d’aller vite afin de permettre l’entrée en vigueur rapide de ce texte très attendu par le monde agricole. Il est très attendu, parce qu’il est absolument essentiel. Dans la gigantesque tectonique des plaques qui s’est engagée dans l’ordre international, le vieux monde se meurt et emporte avec lui toutes nos certitudes : la paix, que d’aucuns croyaient perpétuellement installée en Europe, s’est fracassée sur le mur de la guerre et, tandis que la menace rampe jusqu’à nous, nos alliances d’hier paraissent plus fragiles que jamais. Pourtant, le nouveau monde tarde à apparaître et, dans ce clair obscur où surgissent les monstres, les Français demandent les moyens de parer au vent mauvais qui souffle sur le continent. Alors, mesdames, messieurs les sénateurs, face à cette instabilité qui croît, notre priorité doit être de réancrer la France dans ce qui a été et continuera d’être le socle le plus solide et le plus fidèle de toutes les civilisations de toutes les civilisations humaines : l’agriculture. Pour qu’elle soit tout à la fois notre rempart et notre force face aux menaces qui perlent à l’horizon, il nous la faut souveraine. Aussi, le projet de loi que vous avez désormais la responsabilité de consolider et de voter se doit d’ériger en intérêt général majeur la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture française, de la pêche et de la forêt. Il reconnaît, en outre, l’agriculture comme participant au potentiel économique de la France, constituant ainsi un intérêt fondamental de la Nation. Il ne s’agit pas là de se payer de mots, car ce sont bien les intérêts fondamentaux – oserais je même dire vitaux qui sont en cause lorsqu’il s’agit de garantir la souveraineté alimentaire et agricole. Ces deux avancées majeures permettront, dans tous les débats à venir, que les autorités administratives ainsi que les juges prennent en compte la place particulière de notre agriculture. Aussi est il crucial, au titre I, de doter la politique en faveur de la souveraineté alimentaire de priorités et de finalités solides, ambitieuses et précises. Les débats sur ce point ont été nombreux, les propositions parfois trop bavardes. Nous devons collectivement faire preuve de pragmatisme pour que la politique de souveraineté alimentaire se concrétise avec efficacité. efficacité. L’État doit apporter un soutien ferme à nos filières, notamment les plus exposées, pour les accompagner sur le chemin de la croissance, du progrès et de la vitalité, sur le chemin de l’accroissement du potentiel agricole de notre pays pour nourrir l’ensemble de notre population et pour accroître le rayonnement de nos filières au delà de nos frontières. L’efficacité commande toutefois d’organiser cet effort. La programmation pluriannuelle qui avait été envisagée par l’Assemblée nationale, aussi louable soit elle dans son principe, aurait marché sur les plates bandes du plan national stratégique élaboré dans le cadre de la Elle aurait par ailleurs conduit le Gouvernement à imposer aux filières une direction trop verticale. C’est une ligne rouge. L’avenir de nos filières se construit avant tout par et avec elles. Elles doivent déterminer souverainement leur ambition, car ce sont elles qui connaissent le mieux la réalité du terrain, ses contraintes comme ses opportunités. C’est pourquoi je souhaite que nous fassions le pari de la confiance donnée à la profession à travers l’instauration de conférences de la souveraineté alimentaire. Celles ci confieront aux filières le soin de définir collégialement, avec l’accompagnement de l’État, des objectifs à dix ans pour améliorer de façon substantielle le potentiel agricole de notre nation. Des rapports d’avancement permettront aux pouvoirs publics de suivre l’état de réalisation de ces objectifs et, si nécessaire, de mettre en œuvre des mesures pour les atteindre afin d’assurer la progression de notre souveraineté alimentaire et agricole. C’est toute la portée de ces conférences. Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, face aux périls de l’époque, il faut un changement de cap. C’est désormais l’autonomie stratégique que nous visons. Mesdames, messieurs les sénateurs, une fois jetées les fondations de cette ambition nouvelle, il faut nous saisir à bras le corps de ce qui constitue la clé de voûte de la reconquête de notre souveraineté alimentaire : le renouvellement des générations.

Il faut, là aussi, faire preuve d’ambition. Les objectifs que nous nous fixons dans le présent projet de loi sont clairs : il s’agit notamment d’augmenter de 30 % le nombre d’apprenants dans les filières agricoles et agroalimentaires d’ici à 2030. Le défi est grand, mais pleinement Avant d’en venir au contenu du projet de loi proprement dit, je tiens à souligner dans cet hémicycle que l’atteinte de ces objectifs dépend aussi de nous et du discours que nous véhiculons sur le monde agricole. L’agriculture française fait face à de nombreux défis, existentiels pour certains d’entre eux, personne ne le niera, mais elle n’est pas un champ de ruines pavé de larmes et de misère comme je l’entends dire parfois. Les problèmes existent, il n’est pas question de les nier, nier, mais ce pessimisme effraie et décourage jusqu’à la plus solide des vocations. Pourtant, dans une période où la jeunesse est en demande de sens, les métiers du vivant en sont une source infinie,

Aussi, chacun d’entre nous doit être en mesure de tenir un discours positif sur l’avenir de l’agriculture, pour susciter l’envie, l’engagement.

Vous avez permis, mesdames, messieurs les sénateurs, de franchir une nouvelle étape dans le renforcement de l’attractivité de l’agriculture : un volontariat agricole est désormais créé et je m’en réjouis. Il permettra aux personnes extérieures au milieu agricole de découvrir les métiers du vivant et, nous l’espérons, de susciter des vocations. Cette politique d’attractivité s’accompagnera d’un enrichissement des formations disponibles au sein de l’enseignement agricole. Je pense bien sûr à la création du bachelor agro, dont nous ambitionnons de faire un niveau de formation de référence dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, supérieur (BTS) agricole et le diplôme d’ingénieur. Il était par ailleurs indispensable de compléter les missions assignées à l’enseignement agricole afin de l’adapter aux défis de notre temps.

Les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique ; il est donc primordial que nos établissements agricoles puissent organiser des formations visant plus largement les transitions climatique et environnementale. Le texte que nous avons la responsabilité de voter doit nécessairement les intégrer.

Si, comme je le pense, cette politique de formation nous permet d’augmenter substantiellement le nombre d’agriculteurs en devenir, il nous faut en parallèle renforcer notre politique d’installation et de transmission. De nouveau, plutôt que de faire de grandes phrases, il faut nous fixer des objectifs chiffrés : en 2035, notre pays devra compter 400 000 exploitations et 500 000 exploitants agricoles. dans ce domaine également, notre ambition est grande. L’atteinte de ces objectifs dépend beaucoup de la force de l’accompagnement que l’État sera en mesure d’apporter lors de l’installation ou lors de la transmission des exploitations.

Ce diagnostic va, j’en suis persuadée, devenir un outil incontournable pour les exploitants, notamment dans les périodes clés, au moment de l’installation ou de la transmission. J’ajoute que l’Assemblée nationale a beaucoup enrichi le diagnostic modulaire. diagnostics, les exploitants pourront prendre des décisions éclairées sur le pilotage de leur exploitation et asseoir leur performance économique, sociale et environnementale.

Je regrette là aussi cette nouvelle terminologie, dont nous débattrons. France Services agriculture, je le rappelle, est un intitulé qui parle désormais à nos concitoyens et qui permettra d’attirer réellement de nouvelles personnes vers les métiers Ce guichet unique sera le lieu de maturation des projets, que ce soit pour lancer une activité ou pour la cesser et trouver un repreneur. Mais, mesdames, messieurs les sénateurs, l’ensemble de ces mesures

Aussi, je souhaite mettre un terme à toutes les formes de stigmatisation, voire de criminalisation, de la profession, qui minent terriblement le moral de nos agriculteurs. Les hommes et les femmes pour qui le sens d’une vie est précisément d’être connecté à la nature et à ses cycles ne peuvent décemment pas risquer des poursuites pénales pour des atteintes involontaires à l’environnement, les peines encourues allant jusqu’à l’emprisonnement. Aussi la dépénalisation de ces actes est elle un impératif majeur. Grâce à ce texte, nous substituerons à des sanctions pénales lourdes, résultant d’une surtransposition du droit européen,

Nous devons également poursuivre le travail que j’ai entamé en matière de simplification de la vie des paysans. Car la simplification doit être le maître mot de notre politique agricole à court terme. Il s’agit de faire en sorte que les agriculteurs passent plus de temps dans leur exploitation que devant leur ordinateur. C’est pourquoi nous créerons un régime unique de la haie. La prolifération et la complexité des réglementations en vigueur nuisent à l’objectif de protection de la biodiversité.

c’est aussi réduire les délais des recours contentieux contre les projets agricoles ou les ouvrages hydrauliques, dont les durées de traitement, de plus de cinq ans aujourd’hui, sont une source d’insécurité majeure pour nos agriculteurs.

Enfin, la sécurisation du statut jurisprudentiel du patou est une avancée essentielle pour nos éleveurs, qui doivent lutter au quotidien face à la prédation du loup. Vous avez souhaité enrichir les dispositions sur la protection des troupeaux en y intégrant la reconnaissance de la non protégeabilité de certains troupeaux, notamment bovins et équins.

Nous avions déjà travaillé sur ce point au niveau réglementaire et votre proposition, sur laquelle je reviendrai, car elle suppose des explications juridiques complexes, permettra de sécuriser les arrêtés en préparation.

Sur la réparation, nous avançons aussi : le principe d’indemnisation est acté et les services des ministères de l’écologie et de l’agriculture travaillent à établir les grilles financières d’indemnisation. Le Gouvernement tient donc ses engagements pour accompagner nos éleveurs face à la prédation. Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, avant de conclure, je ne peux pas m’abstenir d’évoquer devant vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur : l’accroissement de la place des femmes en agriculture. Leur engagement dans le monde agricole, aujourd’hui substantiel, n’est pas suffisamment reconnu, alors même que leur place est et sera centrale dans le renouvellement des générations.

du vivant et le sens qu’ils donnent doivent être accessibles à tous, sans distinction de sexe. Cette conception de l’agriculture doit pénétrer tous les esprits. C’est la raison pour laquelle les maîtres de stage et d’apprentissage seront eux aussi sensibilisés à la nécessité de recruter des filles.

Je propose ainsi que l’accès au statut de chef d’exploitation soit facilité, que l’État se dote d’une stratégie pour lever les obstacles de toute nature aux projets d’installation des agricultrices et que le futur réseau France Services agriculture agriculture veille particulièrement à ce que les femmes, qui s’installent plus tard que les hommes, puissent bénéficier dans les faits de programmes d’accompagnement, lesquels facilitent grandement l’installation. Une reconnaissance explicite de leur rôle dans la loi, couplée à une action forte en matière de formation et d’installation : tels sont les outils qui nous permettront d’accroître concrètement la place des femmes en agriculture, mesdames, messieurs les sénateurs. Avec ce texte, nous semons les premières graines de la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Elles germeront, j’en suis convaincue. Cette entreprise immense est une nécessité pour notre pays, elle est tout autant une nécessité humaine. Car en redonnant à notre agriculture la place qui lui est due, ce sont nos agriculteurs qui retrouvent leur rang, leur dignité. Il s’agit là de la seule voie possible pour substituer au vent de colère qui s’est engouffré dans leur cœur un vent d’espoir et de foi retrouvée en l’avenir.

à condition d’avoir une portée juridique. Nous y reviendrons. La logique est la même lorsque nous déclarons que l’agriculture est d’intérêt général majeur et que nous inscrivons dans le code rural un principe de non régression de la souveraineté alimentaire, assorti d’un principe de non surtransposition des règles européennes. Le but

Nous avons essayé – je dis bien : essayé – de rendre cet article plus lisible et moins stigmatisant, et de concrétiser l’objectif de simplification des réglementations applicables aux haies. En la matière, la seule politique qui vaille est celle de la territorialisation : dans certains départements, dont le mien, il n’y a jamais eu autant de haies depuis 1950, que cela plaise ou non. Il suffit de regarder les photos aériennes sur Géoportail, ce que nous pouvons tous faire. Je vous invite Je ne nie pas que, dans d’autres départements, le linéaire a eu tendance à décliner. Veillons donc à protéger les haies quand elles disparaissent, bien sûr, et à laisser les agriculteurs vivre quand ils en sont entourés Avec l’article 17, nous offrons à l’aquaculture française la possibilité de bénéficier des mêmes règles que ses concurrents européens, ni plus ni moins. Je rappelle que nous importons déjà 70 % du poisson que nous consommons.

efforcé en commission de consolider l’enseignement agricole en veillant à placer l’acquisition des compétences au centre des priorités. Sans jeunes formés, compétents et motivés, nous ne pourrons ni assurer le renouvellement des générations ni faire face aux défis économiques et environnementaux de demain. L’Assemblée nationale a déjà renforcé et amélioré plusieurs points clés. Madame la ministre, vous y avez pris part lorsque vous étiez députée. Je pense par exemple à l’article 5 concernant le bachelor agro, dont je soutiens pleinement à la fois le principe et la dénomination. En effet, il faut reconnaître les réalités internationales du marché du travail et l’attrait que peut exercer un tel intitulé. Il faut aussi différencier cette formation des nombreuses licences professionnelles qui existent dans notre pays.

agricole viable, vivable et résiliente. Par ailleurs, je reste très attaché à la diversité de l’enseignement agricole français, qui a toujours comporté

toutes les incitations et toutes les dynamiques positives, notamment la qualité de l’accompagnement, plutôt que les contraintes. Le guichet unique prévu à l’article 10 est une mesure phare destinée à simplifier

: une information pour toutes les personnes intéressées par l’agriculture et un accompagnement uniquement pour celles qui ont un projet formalisé d’installation ou de reprise. Quoi qu’il en soit, il me semble que la priorité doit être de donner envie aux jeunes de s’installer et de rester. Enfin, permettez moi de rappeler que la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, adoptée la semaine dernière par notre assemblée, à mes yeux un complément logique du présent projet de loi d’orientation. Installer des jeunes ne suffira pas si les normes les découragent ou si la rentabilité n’est pas au rendez vous. Je pense fermement que l’attractivité du métier repose avant tout sur des conditions d’exercice équitables, par rapport à nos partenaires européens en particulier, et des conditions d’exercice vivables. C’est pourquoi il nous faut aussi réfléchir à d’autres organisations, notamment à des formes d’installation en commun, plus progressives, auxquelles je tiens beaucoup. Ce texte ne réglera pas tout, madame la ministre, mais il fixe assurément un cap

ans après la loi Rocard, fondatrice de l’enseignement agricole, ce texte ouvre un nouveau chapitre. C’est là une nécessité urgente, tant les chiffres sont vertigineux s’agissant du besoin de renouveler les générations. Laurent Duplomb et Franck Menonville, dont je veux saluer l’excellent travail,

atteignables, selon le ministère, par la mise en œuvre d’un « choc d’attractivité ». Le texte prévoit pour cela d’abord une meilleure articulation entre l’éducation nationale et l’enseignement agricole, car les car les familles comme le corps enseignant ont trop souvent des connaissances assez lacunaires sur les perspectives offertes. Le texte prévoit également une autre innovation : la création d’une cartographie régionale des besoins de consolidation et d’ouverture de sections de formation. Ce dispositif donnera une visibilité pluriannuelle aux classes à faible effectif et devrait leur garantir des moyens supplémentaires en cas d’augmentation significative du nombre d’élèves. Enfin, le texte crée un nouveau diplôme de l’enseignement supérieur court, afin de répondre à un double objectif

Enfin, la commission de la culture souhaite que soit modernisée une procédure disciplinaire devenue obsolète dans l’enseignement supérieur. C’est une demande forte des établissements concernés. nous avons aussi évoqué plusieurs points de vigilance. D’abord, si ce texte se concentre sur la formation dans les domaines agricole et agroalimentaire, n’oublions pas que l’enseignement agricole forme au delà des métiers de l’agriculture. Je pense aux métiers des services à la personne et d’animation des territoires par exemple. Alors, veillons à ce que l’augmentation des moyens alloués aux formations agricoles et agroalimentaires ne se fasse pas au détriment octroyés aux filières des services à la personne et de l’animation des territoires. Les besoins sont très nombreux, particulièrement dans les départements ruraux. Ensuite, nous souhaitons alerter sur les dérives potentielles de l’appellation bachelor agro. Aujourd’hui, dans l’enseignement supérieur, certaines officines privées lucratives jouent sur la confusion entre diplômes et titres. Elles proposent des formations souvent dénommées bachelor, sur la base de titres loués au répertoire national des compétences,

Enfin, les efforts en faveur de l’enseignement agricole seront vains sans amélioration des revenus et des conditions de travail des agriculteurs. À cet égard, la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a toute sa pertinence elle est même, disons le, intrinsèquement liée à ce choc d’attractivité. La

le texte dont nous commençons l’examen a connu un destin contrarié. Mais nous sommes enfin à la dernière étape du marathon législatif, avec la première lecture de ce projet de loi. ces retards est simple : ce texte, attendu par le monde agricole, a été une victime collatérale des soubresauts politiques de l’année 2024, qui ont conduit au report de son examen et à des délais inhabituellement longs – qui nous ont fait relativiser l’efficacité de la procédure accélérée. Ces retards successifs ont désespéré une partie du monde agricole. Ils ont d’ailleurs conduit à une mobilisation inédite des syndicats agricoles pour sortir ce texte de son enlisement législatif. Depuis plus d’un an, ce projet de loi fait en effet miroiter aux agriculteurs et aux paysans des solutions pour les accompagner face aux défis multiformes qu’ils doivent relever déprise rurale, concurrence extérieure, changement climatique, stress hydriques à répétition, évolution des attentes et des préférences des consommateurs, mais également instabilité réglementaire en matière sanitaire et environnementale. Il était temps que le supplice législatif prenne fin et que notre assemblée puisse travailler avec un exécutif prêt à prendre des engagements pérennes, pour donner un cap et des orientations à ce que sera l’agriculture de demain. À l’aune de cette exigence, ce projet de loi est il à la hauteur des défis ? Ses objectifs sont nobles : préparer l’avenir de l’agriculture, assurer le renouvellement des générations et former suffisamment d’actifs agricoles, tout en amorçant une trajectoire d’adaptation pour sortir de l’impasse climatique. Mais il faut se rendre à l’évidence, ce projet de loi ne deviendra aucunement la grande loi d’orientation que nous espérions. Il fut un temps où le législateur était capable de synthétiser les préférences collectives en matière agricole, mais cette époque est manifestement révolue, peut être parce que les représentations sociales de l’agriculture ont changé. Mais ce projet de loi ne doit pas pour autant être jeté aux orties. L’État doit accompagner des modèles agricoles à la croisée des chemins et innover dans son soutien pour faciliter la vie de l’agriculteur et lui faire confiance. La forte demande de simplification répond à une impérieuse nécessité pour ne pas désespérer des acteurs qui font preuve de bon sens et qui ont déjà bien assez à faire, au champ ou à l’étable. Offrir un cadre simplifié d’action, pour libérer l’activité agricole de normes excessivement lourdes ou contradictoires, sans diminuer l’ambition environnementale : voilà le mandat que le monde rural nous confie. La voie est étroite, nous le savons. L’objectif, à mes yeux, est de garantir notre souveraineté agricole et de promouvoir une agriculture compétitive, et économiquement viable. L’agriculture doit être érigée au rang d’intérêt fondamental de la Nation. La souveraineté alimentaire ne se décrète pas : elle se construit en sécurisant nos filières de production, en soutenant nos agriculteurs et en investissant dans une agriculture durable, capable de produire une alimentation saine, sûre et accessible à tous, conformément au principe de souveraineté alimentaire. C’est ce que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’est efforcée de promouvoir. Ce texte est loin d’être parfait. Il a quelque chose d’un fourre tout, reflète de nombreux impensés, comporte des incohérences et des orientations brouillées, à force d’empiler des dispositifs, parfois à la limite du bavardage législatif. Il manque aussi d’ambition pour renforcer la durabilité des productions alimentaires. Aucun mécanisme n’est élaboré pour protéger les agriculteurs de la concurrence déloyale et des défaillances de marché. N’attendons donc pas de ce projet de loi qu’il résolve tous les problèmes ou qu’il fixe de façon intangible le cadre optimal pour accompagner les agriculteurs face aux défis. Il ne fera certainement pas date et il ne pourra que décevoir ceux qui placent de trop grandes attentes dans un texte finalement plus de circonstance que d’orientation. Cependant, malgré ses défauts et ses lacunes, ce projet de loi apporte des évolutions bienvenues et nécessaires, tout en ayant le mérite de traiter de sujets qui concernent l’activité quotidienne des agriculteurs. Il pose les bonnes questions, même s’il apporte rarement les bonnes réponses. En l’état, il est cependant de notre devoir d’apporter une partie des évolutions attendues par la profession agricole et d’imaginer des dispositifs pour limiter l’insécurité juridique qui entoure certains projets agricoles.

Le renouvellement des générations en agriculture impose de répondre à la question suivante : quel avenir souhaitons nous pour l’enseignement agricole, qui forme nos agriculteurs de demain, et qui est fondamental dans la transmission des exploitations ? La mission d’information sur l’enseignement agricole, que Jean Marc Boyer avait menée avec la sénatrice Nathalie Delattre en 2021, avait conclu à l’urgence d’une transition agropolitique afin de donner une stratégie et des objectifs clairs à l’enseignement agricole. Or la mobilisation des agriculteurs – et en particulier des jeunes agriculteurs – ces derniers mois a bousculé quelques fondamentaux. Certes, les missions essentielles confiées à l’enseignement agricole restent la base d’un enseignement innovant et performant avec une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue, une animation de développement des territoires, une insertion sociale, scolaire et professionnelle, le développement, l’expérimentation et l’innovation, des actions de coopération internationale. Mais il s’avère aujourd’hui nécessaire de traiter deux enjeux majeurs de développement des filières de production : la transformation agricole, qui allie performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, et le développement de modèles économiques agricoles adaptés à chaque région, prenant en compte les conditions géographiques et climatiques, notamment en zone de montagne. Le réseau de l’enseignement agricole, avec ses 825 établissements, est indispensable pour répondre au défi d’une transition agropolitique et du renouvellement des générations d’agriculteurs. L’enseignement agricole doit regagner ses lettres de noblesse. Il s’est trouvé modifié et dogmatisé vers les filières environnementalistes, et en décalage avec une partie de la profession agricole. Il doit rester ouvert à tous à tous les types d’agriculture. Il y a vingt ou trente ans, 80 % des élèves étaient d’origine rurale et agricole. Aujourd’hui ils ne sont plus que 30 %, et les 70 % restants sont sensibilisés aux notions agricoles, mais pas aux milieux agricoles et à leur environnement naturel. Nos élèves agricoles sont formés pour être des jardiniers de la nature, ce qui ne leur offre pas de réels débouchés. Beaucoup s’orientent donc vers des filières vertes et non plus vers l’élevage ou l’agriculture qualifiée de conventionnelle, qui, pourtant, reste très présente

Cet agri porte un vrai préjudice à la profession agricole, ainsi stigmatisée. L’enseignement agricole a su montrer ses facultés d’adaptation à l’évolution de l’agriculture et à sa modernisation tout au long du XX siècle. Il a su évoluer avec la révolution technique et la mécanisation. Aussi, tous les moyens de communication, d’information et d’orientation doivent ils être mis en œuvre pour sensibiliser les parents, les enseignants, les collégiens, les lycéens. Pour cela, j’approuve la proposition de la nomination dans chaque département d’un correspondant pour l’enseignement agricole. L’enseignement agricole doit retrouver son essence et permettre l’installation de jeunes agriculteurs pour toutes les agricultures, de la viticulture à la production laitière, fromagère, bovine, ovine. La lutte contre les stéréotypes de genre doit permettre de donner aux filles et aux femmes toute leur place et favoriser un accès diversifié à l’enseignement supérieur agricole. Dès lors que la souveraineté alimentaire redevient une priorité politique, l’enseignement agricole doit permettre aux nouveaux agriculteurs qui s’installent de bâtir un projet économique et entrepreneurial viable, en s’adaptant aux nécessités de la transition agronomique et climatique, aux attentes du citoyen et du consommateur. Il doit aussi intégrer une ruralité vivante, dynamique et porteuse de projets. Il importe enfin de lutter contre la désertification vétérinaire dans les territoires ruraux et de mobiliser l’enseignement agricole sur l’enjeu du bien être de l’agriculteur, ses conditions de travail et sa rémunération, problématiques majeures. Nous devons aussi renforcer l’attractivité de l’enseignement, avec une attention accrue aux enjeux de desserte et de conditions d’accueil des apprenants. La parole

XXI siècle. Avec ce projet de loi, dont la fermentation a été exceptionnellement longue, nous voulons voter du concret pour changer leur vie ; voter pour affirmer le caractère d’intérêt général majeur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture voter pour créer des outils qui formeront les nouvelles générations d’agriculteurs ; voter pour faciliter les transmissions et les installations, notamment d’un point de vue financier voter pour leur simplifier la vie ; voter, enfin, pour renforcer la préservation de notre environnement, car c’est en agissant ainsi que nous protégerons nos agriculteurs des conséquences déjà dramatiques du dérèglement climatique. Mes chers collègues, tous ces enjeux sont cruciaux et j’espère que nos débats permettront d’enrichir, une fois de plus, les mesures contenues dans ce texte. En premier lieu, garantir notre souveraineté alimentaire dans les années à venir exige de notre part, en tant que législateur, d’affirmer juridiquement le caractère d’intérêt général majeur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Affirmer cela, c’est influencer pour l’avenir les politiques publiques qui seront menées par le Gouvernement et envoyer un signal clair pour les prochains contentieux concernant ces activités. Évidemment, il ne s’agit pas de placer l’agriculture au dessus de l’environnement, mais de mieux équilibrer la balance. Le deuxième sujet majeur, c’est la formation. Comment pourrons nous être souverains demain si nous ne formons pas davantage d’agricultrices et d’agriculteurs ?

Face au défi du renouvellement des générations, ce projet de loi apporte des réponses concrètes et utiles. Je pense à la création du bachelor agro, qui sera reconnu comme un Le groupe RDPI proposera d’ailleurs, au cours des débats, de préciser le contenu des enseignements de cette formation, afin qu’elle prenne en compte les enjeux agricoles des territoires ultramarins. Je pense aussi à la création du contrat territorial de consolidation ou de création de formations, qui permettra d’augmenter le nombre de jeunes formés par la voie initiale scolaire dans les établissements de l’enseignement agricole technique. Mais, si nous voulons attirer davantage de jeunes agriculteurs, nous devons également penser à l’attractivité financière. De ce point de vue, l’aide au démarrage prévue dans le texte pour les nouveaux professionnels sera la bienvenue. de même de l’expérimentation, pendant trois ans, d’une option intitulée « Écologie, agronomie, territoires et développement durable » pour quelques élèves de seconde dans notre pays. Je ne doute pas que cette option suscitera la curiosité, et peut être même des vocations. Toutes ces solutions seront utiles pour sensibiliser les jeunes générations et former les nombreux professionnels dont nous aurons besoin pour être souverains.

Qu’il s’agisse de la création du réseau France Services agriculture, qui peut être un véritable levier pour aider nos agriculteurs à transmettre leurs exploitations et à préparer la suite, ou de la mise en place d’un droit à l’erreur pour les agriculteurs, nous avons l’occasion, neuf mois après la présentation de ce texte en Conseil des ministres, de débattre et de voter des mesures pour simplifier la vie des professions agricoles. Lorsqu’on parle de simplification, je pense aussi aux chiens de protection de troupeaux et à la responsabilité pénale de leurs propriétaires, que nous aborderons également dans nos débats. Notre groupe proposera d’élargir la non protégeabilité aux troupeaux caprins face aux attaques de prédateurs comme les loups

Cela permettra de clarifier les choses pour nos agriculteurs, avec une définition claire et une stratégie nationale. Mes chers collègues, à nous de saisir cette occasion pour répondre aux agriculteurs, pour les rassurer et voter une loi d’orientation pour l’avenir de notre agriculture, véritable symbole d’un message de confiance et de soutien envers celles et ceux qui travaillent pour nous nourrir.

Entre les paysans et notre pays, le lien s’est déchiré. Remplacé, trop souvent, par un nauséabond mélange de nostalgie, de mépris et d’accusations. Il est temps, plus que temps, de retisser. » Ensemble, retissons

un jour, peut être, nous examinerons un texte sur l’avenir de notre agriculture qui pense vraiment l’avenir de cette profession dans sa globalité. Un jour, peut être, mais pas aujourd’hui Les textes se suivent, et toujours aussi peu de transversalité… Pourtant, dans nos exploitations, dans nos fermes, les enjeux pour l’avenir de nos entreprises, nous les connaissons. Il y a le revenu, avec l’analyse des coûts de production, le marketing, les marchés, la vente, le foncier, etc. Il y a la diversification

Initialement conçu pour relever les défis liés à la préservation de notre souveraineté alimentaire, ébranlée par le dérèglement climatique et la crise des vocations, ce projet de loi incarne désormais la réponse de l’exécutif à la colère de nos agriculteurs, en attente de mesures concrètes simplifiant, valorisant et sécurisant l’exercice de leur activité. Il faudrait par exemple changer de paradigme, et faire en sorte que les services de l’État mettent fin à la suspicion, qu’ils soient davantage dans leur rôle d’accompagnement et de conseil. La confiance, j’en suis sûr, peut régler beaucoup de maux. Ce texte s’est éloigné d’un de ses objectifs initiaux, à savoir rebâtir notre souveraineté alimentaire en répondant notamment aux défis du changement climatique.

Je pense notamment à ce que l’on appelle les aménités environnementales. Il faut développer les paiements pour services environnementaux territoriaux, qui peuvent apporter des revenus pour les services induits, comme la lutte contre les incendies ou les inondations. Les Les agriculteurs maintiennent les milieux ouverts, ils entretiennent nos paysages, que les urbains savent apprécier le week end sans avoir conscience du travail que font ceux ci sur leur environnement. L’agriculture est l’un des secteurs d’activité les plus sensibles à l’évolution du climat et les plus dépendants du fonctionnement des écosystèmes. L’objectif d’une agriculture économiquement et écologiquement viable, rémunératrice, diversifiée, durable, répartie sur l’ensemble du territoire, doit prédominer et servir de mise en garde contre la stérilité de l’opposition entre modèles agricoles. Je l’ai encore dit la semaine dernière : nous avons tout à perdre à faire de la politique sur le dos de nos paysans.

Ces mêmes collègues savent hurler contre les surtranspositions, mais composent en en acceptant certaines pour aller dans le sens du vent. Il y a un parti pris en faveur de la compétitivité, au détriment de l’environnement et de nos ressources. C’est dommage Face au déclin de notre agriculture, l’urgence d’un sursaut est nécessaire, dans un équilibre constructif. Que faire, donc ? Le RDSE a voulu, une fois encore, que l’agriculture soit cause nationale. proposition du rapport intitulé, que j’ai rédigé avec notre ancienne collègue Françoise Férat en 2021. Plus qu’un symbole… Ce projet de loi reflète la consécration d’une programmation pluriannuelle de l’agriculture. ci devra être établie avant le 1 juillet 2025, puis tous les dix ans, et définir les modalités d’action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l’Union européenne. Elle précisera en outre, par filière, des objectifs nationaux de production compatibles avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie bas carbone et la stratégie nationale pour la biodiversité. Je m’en réjouis.

si l’on fait preuve d’honnêteté, on sait que tous les agriculteurs n’auront pas l’irrigation. Mais la reconstitution des sols de manière durable donne de meilleurs rendements, tout autant qu’une rétention d’eau et une capture de carbone. Il faut le dire. Avec quels moyens, ? Une programmation sans budget, c’est une parole sans actes. Et les coupes sombres de dernière minute au projet de loi de finances ne nous ont pas rassurés. Madame la ministre, même en étant le plus optimiste possible,

Mais pensez vous honnêtement qu’il faille privilégier la formation et la transmission alors qu’aucun levier pour l’attractivité n’est actionné ? Qu’est ce qui va motiver un agriculteur à transmettre son outil à ses enfants ? Il s’agit de son objectif premier et de sa plus grande fierté. Mais s’il sait que cela va être la galère, il ne fera pas le choix de transmettre. Qu’est ce qui va motiver un jeune à devenir agriculteur ? C’est à ces questions qu’il fallait répondre.

Nous avons ensemble, tous ensemble, l’ambition de répondre au malaise agricole, alors que près de 40 % d’entre eux évoquent un sentiment d’abandon et un système à bout. Pour cela, le bon sens paysan, fait de sens pratique et de la capacité à résoudre les problèmes de manière simple, pratique et efficace, peut inspirer un. Les mots

sur vingt quatre, où femmes, hommes, conjoints, enfants vivent l’exploitation au quotidien. La main d’œuvre familiale ne doit donc pas être considérée comme du travail dissimulé. L’entraide rurale n’est pas du travail au noir. Il faut plus de souplesse dans la gestion de la main d’œuvre. Dans les régions transfrontalières comme la mienne, la distorsion de concurrence est aussi une réalité vécue au quotidien. Alors, revenons au bon sens paysan, encore lui, et appliquons tout simplement les mêmes règles à tous ceux qui vendent les produits agricoles sur notre territoire. Ce n’est pas le cas Au nom de quel paradoxe peut on exiger de nos producteurs l’exemplarité sanitaire et environnementale, tout en nous montrant laxistes pour les produits que nous importons ? importons ? Dans ma région, on produit notamment de la betterave à sucre. Comment expliquer à mes agriculteurs – et aux agriculteurs français en général – que les producteurs ukrainiens ont toujours accès huit matières actives interdites chez nous, mais qui sont transformées sans contrainte et qui continuent à être distribuées par les industries agroalimentaires ? Il faut donc poursuivre et intensifier le travail sur les clauses miroirs. Le foncier est aussi un enjeu déterminant. Trop souvent, dans ma région, la spéculation foncière pénalise nos exploitants, qui doivent faire face à la pression des agriculteurs belges. Il faut de nouveau remettre l’ouvrage sur le métier, notamment avec les rural (Safer). La simplification administrative sera au cœur de nos débats. Là encore, le bon sens paysan, toujours lui, doit nous animer plus que jamais. Soyons pragmatiques et travaillons en confiance. Hélas ! hélas ! trois fois hélas ! la complexité administrative alourdit notre quotidien et nuit à la rentabilité de nos exploitations. Je prendrai l’irrigation. On impose à nos agriculteurs de noter jour par jour l’eau consommée, alors que nos dispositifs de pompage sont équipés de compteurs. Pourquoi ne pas simplement relever ces compteurs avant et après la saison, pour connaître précisément la consommation ? Ces contrôles excessifs sont inutiles et doivent être simplifiés. Même remarque sur la PAC : les aides sont devenues un labyrinthe bureaucratique. Par exemple, la valeur des points d’écorégime est totalement déconnectée du terrain. La betterave et la pomme de terre, particulièrement cultivées dans mon département, sont considérées comme une seule et même culture. Pourtant, je mets au défi quiconque de faire des frites avec des betteraves ou du sucre avec des pommes de terre Il est urgent d’adapter les critères aux réalités agricoles. Ce projet de loi d’orientation agricole arrive enfin au bout de son parcours. En l’adoptant, comme nous l’espérons, le Sénat enverra un signal positif à nos agriculteurs. Ils l’attendent depuis huit mois. Ce n’est pas encore une loi cadre, mais, même s’il reste beaucoup à faire pour en faire une vraie orientation, une ambition, elle est nécessaire. Vous pourrez compter sur les élus du groupe Union Centriste pour faciliter la vie de celles et de ceux qui nous nourrissent. Mes chers